ainsi l'autorisation parlementaire. Ce choix implique aussi, à nos yeux, l'absence de dispositions fiscales dans les textes de fin de gestion, qui participe aussi à la stabilité fiscale pour les entreprises comme pour les ménages. comme pour les ménages. La fin de gestion prend cette année, vous le constatez, une forme particulière, pour ne pas dire extraordinaire, compte tenu de la nécessité de recharger les dispositifs d'urgence pour faire face à l'évolution de la pandémie et financer de nouvelles mesures de soutien. Notre responsabilité est d'assurer le financement de ces dispositifs de soutien aux entreprises et aux Français, et de tenir compte de la reprise épidémique à laquelle nous faisons face. Le contexte macroéconomique de cette fin d'année, bouleversé par la seconde vague épidémique, conduit à dégrader les prévisions de finances publiques que nous avions faites pour 2020 au moment de la présentation en conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2021 Lors de la présentation du PLF 2021, nous avions fait preuve de prudence, au vu des incertitudes entourant la situation sanitaire : nous estimions la récession en 2020 à-10 %, alors que la plupart des prévisionnistes la situaient autour de-9 %. Le Haut Conseil des finances publiques avait d'ailleurs souligné cette prudence. La seconde vague épidémique que nous subissons aujourd'hui nous a conduits à dégrader nos prévisions macroéconomiques et nos prévisions de finances publiques pour 2020. Toutefois, cette dégradation reste limitée, à 1 point de PIB, soit une récession de 11 %.

par mois : 6 milliards d'euros pour le fonds de solidarité, 7 milliards d'euros au titre de l'activité partielle, 1 milliard d'euros liés aux exonérations de charges et 1 milliard d'euros au titre du crédit d'impôt pour les bailleurs.

Chacun le sait très bien : la durée et l'intensité des mesures sanitaires au cours du mois de décembre dépendront de l'évolution de la situation épidémique et de l'efficacité des mesures prises depuis quinze jours. jours. Face aux incertitudes sur ces évolutions, nous voulons simplement être en mesure d'aider et de soutenir nos entreprises jusqu'à la fin de l'année, y compris en phase transitoire de déconfinement et y compris si la pire des hypothèses devait se réaliser, ce que, bien sûr, nul ne souhaite. l'expérience de la première vague montre que les mesures d'aide sont ajustées progressivement, et non le jour même du déconfinement, ce qui renforce notre prudence. Au bout du compte, avec ce PLFR 4, nos finances publiques s'alourdissent de plus de 20 milliards d'euros

Certaines mesures d'urgence sont inscrites dans d'autres missions. C'est le cas des aides exceptionnelles de solidarité, pour 1,1 milliard d'euros, qui font l'objet d'ouvertures de crédits au titre de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances

110 millions pour le sport et plus de 50 millions d'euros pour le ministère de l'enseignement supérieur. Je me dois aussi d'informer votre assemblée que le Gouvernement est sur le point de

de la même mission, l'Assemblée nationale a tiré les conséquences de la dynamique constatée des plans de soutien aux filières aéronautique et automobile et des aides à la relocalisation des secteurs critiques. Les députés ont ouvert 82 millions d'euros pour 2020 à ce titre. Ces fonds correspondent à des anticipations de versements au titre de ces dispositifs, inscrits dans le plan de relance,

Conscients de l'appréhension des EPCI en ce qui concerne leur capacité d'autofinancement en 2021 et 2022, nous proposerons que ces avances remboursables soient, à titre exceptionnel, imputées en section de fonctionnement et remboursées entre 2023 et 2027, pour laisser aux collectivités territoriales le temps de retrouver une situation financière satisfaisante.

visant à rétablir l'ancien dispositif du droit à l'image collective, appliqué entre 2004 et 2010, contre l'avis du rapporteur général et du Gouvernement. Le Gouvernement reste opposé à ce dispositif, pour des raisons tant de forme que de fond.

Ainsi, le bénéfice de ce dispositif n'était nullement lié, en pratique, aux revenus réellement perçus au titre de l'exploitation du droit à l'image. Par ailleurs, la baisse de cotisations sociales était très largement concentrée sur quelques clubs de sport professionnel, aux ressources les plus importantes. Enfin, aucun impact sur la compétitivité des clubs n'avait pu être véritablement observé. Il est toutefois possible que le nouveau dispositif soulève des questions dans le cadre de sa mise en oeuvre, même s'il n'est applicable que depuis très récemment. J'entends ces inquiétudes. C'est pourquoi je proposerai qu'un travail soit engagé entre les services de mon ministère, ceux du ministère des sports et le Parlement pour expertiser les éventuelles limites du dispositif actuel et ses améliorations possibles.

Ces chiffres sont porteurs d'espoir : ils démontrent la capacité de rebond de notre économie et la pertinence des outils de soutien que nous avons mis en place. Quand l'économie repart, les recettes publiques repartent aussi. La dynamique constatée sur ce plan nous a permis d'enregistrer un niveau de recettes supérieur à ce que nous attendions, y compris dans la dernière prévision du PLF 2021, présentée au début de septembre.

Le rebond de l'activité au troisième trimestre explique évidemment ces rebonds de TVA et d'IS. En outre, au regard des remontées comptables à fin septembre, les recettes d'impôt sur le revenu sont revues à la hausse de 600 millions d'euros, en raison de revenus des ménages sous-jacents plus élevés que prévu.

Hors mesures d'urgence liées à la seconde vague épidémique, ce projet de loi de finances rectificative comporte un schéma de fin de gestion équilibré entre ouvertures et annulations de crédits. Le niveau des ouvertures et des annulations s'établit à 4,1 milliards d'euros. Les principales ouvertures concernent : le financement des aides personnalisées au logement (APL), pour 1,9 milliard d'euros, du fait principalement du report de la réforme APL en temps réel, mais aussi d'une tendance à la hausse liée à la crise économique

Quant aux annulations, elles portent essentiellement sur les crédits mis en réserve, pour 1,4 milliard d'euros, et sur des crédits sous-consommés du fait de la crise sanitaire. Nous constatons en effet des sous-exécutions pour certaines dépenses immobilières, comme celles du programme de rénovation des cités administratives, mais aussi pour des projets informatiques financés par le fonds de transformation ou pour la sinistralité des dispositifs de garantie créés pour répondre à la crise sanitaire. Le PLFR 4 matérialise aussi notre action de sincérisation du schéma d'emplois.

Par ailleurs, les effectifs augmentent cette année au sein du ministère de la justice, puisque nous avons autorisé des créations de poste en gestion pour rattraper le retard pris dans le traitement des affaires judiciaires et mettre en oeuvre la justice de proximité.

C'est pourquoi, comme je l'ai déjà annoncé à votre commission, je considère que le moment est venu d'engager une réflexion de fond sur le redressement des comptes publics à moyen terme. À cette fin, nous devons travailler sur des scénarios possibles de redressement des finances publiques à moyen terme et moderniser les outils de pilotage des finances publiques, pour renforcer notre capacité à conduire ce redressement en sortie de crise. nous devons travailler à identifier des règles et des modalités de pilotage qui permettraient d'éviter l'accumulation de déficits et de rendre les choix collectifs plus lisibles ; à définir une stratégie de gestion de la dette résultant de la covid et des modalités qui permettraient ; à mieux concilier le principe d'annualité budgétaire et la vision pluriannuelle nécessaire tant pour les ministères en charge des comptes que pour les gestionnaires ; à améliorer les processus d'élaboration et d'exécution des budgets de l'État et de la sécurité sociale, notamment à l'échelon déconcentré ; enfin, à améliorer les outils à la disposition du Parlement.

Nous aurons à fixer l'horizon du remboursement de la dette, du redressement progressif des finances publiques et, surtout, du retour à la croissance, qui rendra les deux premiers objectifs possibles.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis d'un quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ; nous espérons qu'il sera le dernier. Celui-ci est habituel, puisque, à chaque fin d'exercice, un projet de loi de finances rectificative doit tirer les conséquences de l'année écoulée et proposer un schéma de fin de gestion. Ce texte devait donc initialement se limiter à des ajustements budgétaires d'ampleur modeste, même si la fin de gestion se trouve pour le moins perturbée par les événements de l'année.

Ainsi, le Gouvernement a dû revoir à la baisse sa prévision de croissance pour 2020, qui me paraît prudente. Alors que le PLF 2021 tablait sur une chute du PIB de 10 % à l'issue de l'exercice 2020, celle-ci atteindrait finalement 11 %. Ce scénario se fonde sur l'hypothèse d'une perte d'activité de 20 % en novembre par rapport au niveau d'avant la crise, contre 30 % en avril, lors du premier confinement. En réalité, cette hypothèse est sans doute un peu pessimiste. Les premières analyses des instituts de conjoncture tablaient plutôt sur une perte d'activité de 15 la première estimation réalisée par la Banque de France sur une étude conduite auprès des chefs d'entreprise après le confinement confirme ce constat

était attendu, la perte serait très concentrée sur les services marchands, tandis que l'agriculture, l'industrie et la construction seraient relativement préservées. De fait, ces secteurs parviennent à poursuivre leur activité du fait à la fois des modalités plus souples du nouveau confinement, de l'expérience acquise par les entreprises et de la disponibilité des matériels de protection. En tout état de cause, la prévision de croissance gouvernementale est très prudente, tout en incluant déjà une prolongation du reconfinement en décembre.

D'ailleurs, la révision à la baisse de l'hypothèse de croissance n'a pas conduit le Gouvernement à diminuer sa prévision de recettes, laquelle est même, comme le ministre l'a souligné, très légèrement réévaluée par rapport au projet de loi de finances pour 2021, à hauteur de 700 millions d'euros supplémentaires. Ainsi, c'est uniquement la hausse des dépenses liées aux mesures de soutien qui explique la dégradation de la trajectoire budgétaire. Comme vous le savez, ce renforcement porte prioritairement sur les mesures permettant de compenser directement les pertes des entreprises. C'est le cas du fonds de solidarité, dont les crédits augmentent de 10,9 milliards d'euros, des nouvelles exonérations de cotisations sociales, pour 3 milliards d'euros supplémentaires, et de l'enveloppe complémentaire de 3,2 milliards d'euros pour le

Inévitablement, la prévision de déficit pour l'État plonge également, pour atteindre 222,9 milliards d'euros, soit quasiment le niveau prévu l'été Les recettes fiscales ne sont pas en cause pour expliquer ce résultat. Au contraire, après des encaissements plus élevés que prévu au cours de l'été, les estimations de recettes fiscales nettes sont encore réévaluées par rapport à septembre C'est donc, là encore, du côté des dépenses que se trouve l'explication du déficit. En effet, compte tenu de la seconde vague de l'épidémie et du reconfinement, une augmentation de 27 milliards d'euros du niveau des dépenses prévisionnelles de la mission « Plan d'urgence est prévue dans ce projet de loi de finances rectificative. Alors que la prévision de déficit de septembre se fondait sur une hypothèse de sous-consommation de 10 milliards d'euros environ des crédits du plan d'urgence,

Si ces crédits étaient vraiment consommés jusqu'à la fin de l'année, cela nous conduirait à dépenser beaucoup plus pendant les derniers mois de l'année que pendant le premier confinement. Ainsi, le fonds de solidarité disposera de plus de 13 milliards d'euros pour les trois derniers mois de 2020, soit le double des crédits consommés jusqu'à présent. Vous faites donc le choix de la prudence, monsieur le ministre. Votre budget rectificatif repose sur des hypothèses extrêmement conservatoires ; le déficit prévu ne devrait pas être réellement atteint. Des crédits budgétaires pourront probablement être reportés sur 2021- nous en reparlerons dans les prochains jours. D'ailleurs, nous savons déjà que la moitié de l'enveloppe de 20 milliards d'euros prévue au titre du renforcement exceptionnel des participations financières de l'État sera reportée sur 2021. Toujours est-il que, au total, les ouvertures de crédits au fil des quatre lois de finances rectificatives de 2020 sont dix fois plus élevées que les années précédentes.

Outre les nouvelles enveloppes ouvertes au titre des mesures relevant de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », que je viens d'évoquer, les principales ouvertures et annulations de crédits des autres missions du budget de l'État sont souvent, elles aussi, en lien avec la crise c'est, par exemple, le cas de l'ouverture de crédits pour l'aide exceptionnelle de solidarité- un milliard d'euros -ou du financement de la prime à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans- un milliard d'euros en autorisations d'engagement. d'engagement. Les annulations de crédits sont mineures par rapport aux ouvertures mais d'un montant plus élevé que les années normales, la crise ayant assurément différé la réalisation de projets d'investissement, dans des proportions toutefois difficiles à établir. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission des finances ne voit pas davantage de raisons de s'opposer à ce projet de loi de finances rectificative qu'aux trois premiers, sous réserve de quelques ajustements dont je ne dirai que deux mots car nous aurons l'occasion d'en débattre lors de l'examen des amendements.

avons toutefois quelques points de vigilance, monsieur le ministre. Le premier est le fonds de solidarité. Nous regrettons que sa lisibilité initiale ait fait place à une très grande complexité. Par

Nous en sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il convient de prévoir, au-delà de l'aide de 1 500 euros, un renforcement du fonds de solidarité afin de tenir compte des charges fixes de ces structures. Soutenir ces entrepreneurs qui souffrent, c'est assurer une relance plus rapide et efficace demain. Nous devons aider davantage les travailleurs indépendants, qui, ayant investi pour respecter les mesures de protection et de prévention préconisées, ne peuvent donc voir leur activité prendre fin dans ces conditions. Le deuxième point de vigilance est la compensation des pertes de recettes des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Ce sujet, très technique, inclut la question cruciale de l'avenir de nos transports publics. Parmi les comptes spéciaux, deux nouveaux programmes d'avances remboursables sont créés afin de soutenir Île-de-France Mobilités, à hauteur de 1,2 milliard d'euros

en particulier, en inscrivant dans la loi une clause de retour à meilleure fortune, qui assure que les AOM n'auront à les rembourser qu'à partir du moment où elles auront retrouvé un équilibre financier.

Enfin, lors de l'examen du présent PLFR, l'Assemblée nationale a inséré un article additionnel qui prévoit la réintroduction du mécanisme du droit à l'image collective applicable aux sportifs professionnels tel qu'il existait avant 2010. La commission des finances vous propose de supprimer Sur le fond, il y aurait beaucoup à dire sur ce dispositif et les difficultés auxquelles il vise à remédier, mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un sujet de PLFR de fin de gestion et cela n'a pas non plus de lien avec les mesures d'urgence que porte le présent En revanche, nous sommes pleinement conscients des difficultés que rencontre le milieu sportif dans le contexte actuel. C'est pourquoi la commission des finances vous proposera un amendement tendant à revenir sur l'annulation des crédits mis en réserve. Avec ce texte, aujourd'hui, nous traitons la fin de gestion pour l'année 2020 et les mesures d'urgence indispensables pour soutenir notre économie et nos concitoyens. Dans quelques jours, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouverons pour aborder l'examen du projet de loi de finances pour 2021.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi un quatrième projet de loi de finances rectificative. Il faut remonter aux années 2010 et 2011, en pleine crise des dettes souveraines, pour retrouver un rythme aussi soutenu de correction budgétaire.

Compte tenu du deuxième confinement décidé par le Gouvernement, notre pays pourrait connaître une récession de 11 % cette année, une chute inédite depuis 1944. Du fait de la baisse des recettes fiscales et des mesures indispensables de soutien public, le déficit atteindrait 11,3 % du PIB, et la dette publique serait portée à près de 120 % du PIB. Ce dernier PLFR n'est évidemment pas un simple collectif de fin de gestion : il a pour objet de porter les crédits nécessaires pour faire face à l'urgence économique et sociale, et ajoute à ce titre près de 21 milliards d'euros-dont la moitié pour

Pour répondre à cette urgence et débloquer les crédits rapidement, l'Assemblée nationale a d'ailleurs examiné ce texte dans des conditions très contraintes, siégeant jusqu'au petit matin mercredi dernier, ce qui nous permet d'en débattre aujourd'hui ; je tiens à en remercier nos collègues députés. Le Sénat a adopté chacun des trois premiers collectifs budgétaires ; il adoptera sans doute le quatrième. Cependant, la crise ne s'arrêtera pas au 31 décembre de cette année. Non seulement des mesures restrictives pourraient se prolonger- nous ne le souhaitons pas -mais, plus grave, nous commençons à peine à percevoir les répercussions concrètes de la crise, avec son cortège de fermetures d'entreprise et de licenciements qui se traduisent par une forte montée de la précarité. Les réponses à apporter ne sauraient être que ponctuelles, sous la forme d'aides temporaires ou exceptionnelles, ou encore d'avances remboursables, alors que la crise sera sans doute durable. L'idée d'un rebond permettant de retrouver rapidement la situation d'avant-crise n'est pas tout à fait réaliste. Des secteurs entiers sont sinistrés et de très nombreuses famillessont dans des situations très difficiles. Lorsque le plan de relance nous a été présenté au début du mois de septembre pour être intégré au projet de loi de finances, le Gouvernement espérait un redémarrage de l'économie après une activité estivale tout à fait encourageante. Cette dynamique s'est heurtée de plein fouet à la deuxième vague de l'épidémie et au deuxième confinement, qui, pour être moins strict que le premier, se répercute sur le commerce, mais aussi- il faut le dire -sur le moral de l'ensemble des ménages et des acteurs économiques.

Je souhaite que vous nous indiquiez comment vous entendez prendre en compte ces nouvelles données, notamment macroéconomiques. Le projet de budget qui nous est soumis ne doit-il pas faire l'objet, à l'ouverture de nos débats ce jeudi, d'une réactualisation dans toutes ses composantes- équilibre général, recettes, dépenses, notamment d'urgence

Enfin, au-delà du soutien aux entreprises et à l'emploi, quelles mesures structurelles le Gouvernement entend-il prendre pour soutenir, sur le long terme, nos concitoyens les plus fragiles, plus particulièrement la jeunesse, qui, vous le savez, voit son

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en cette quatrième modification de notre budget 2020, je souhaite soulever deux interrogations majeures. Tout d'abord, pourquoi sommes-nous confrontés à une telle calamité économique ? Les difficultés de notre pays, qui étaient déjà grandes avant la crise sanitaire, ont été amplifiées par votre gestion hasardeuse et, même, ruineuse de la crise Votre décision de fermeture de nos commerces de proximité, des cafés, hôtels et restaurants, du monde du sport et de la culture est autant d'huile versée sur le feu d'une crise économique qui se développe chaque jour un peu plus. Tous ces commerçants en phase avec la réalité du terrain étaient pourtant les premiers à appliquer un protocole sanitaire strict et à faire des propositions pour le renforcer. Comme à votre habitude, vous ne les avez pas écoutés. L'exécutif a décidé seul de ce qui est essentiel ou non essentiel, ce qui se traduit, sur le terrain, par des situations d'une stupidité sans nom et par des drames économiques annonçant pour demain de véritables drames humains. Les élus locaux et les corps intermédiaires- syndicats, chambres de métiers et de l'artisanat, chambres de commerce et d'industrie -avaient pourtant formulé des propositions alliant protection sanitaire et protection économique, l'une ne pouvant aller sans l'autre. Plutôt que la concertation, vous avez préféré l'incarcération. Pour une continuité de l'activité dans tous les secteurs économiques, on aurait dû penser un protocole sanitaire composé d'une base minimale stricte puis complété par des adaptations en fonction des territoires et des secteurs d'activité. Mais, pour cela, il aurait fallu que le Gouvernement ne soit pas réfractaire au changement et qu'il daigne traverser la rue pour écouter les maires, les commerçants, les indépendants- ceux qui, jusqu'alors, avaient encore un boulot. Votre fainéantise va nous coûter un pognon de dingue du couvre-feu dans les Bouches-du-Rhône, nous avons essayé de vous alerter par tous les moyens sur le fait que vos mesures étaient administrativement trop compliquées, bêtement unilatérales et globalistes. Nous aurions parlé à un sourd qu'il nous aurait mieux entendus La deuxième inquiétude majeure porte sur les conséquences de vos choix. Qui va payer la faramineuse facture de votre impréparation et de votre incompétence appelées « confinement » Notre endettement est colossal, monsieur le ministre. L'exécutif creuse à la pelleteuse un trou financier pour combler le précédent : c'est le sapeur Camember en habit de président ! C'est de plus inefficace, car cela reste largement insuffisant : les aides promises aux commerçants au mois de juin sont perçues aujourd'hui seulement ; elles ne permettent même pas de payer les loyers. Cerise sur le gâteau, cet endettement massif menace la zone euro d'effondrement. Avec un PIB à-11 % en 2020 et une prévision de-10 % en 2021, ce n'est pas la croissance qui allégera la dette ; ce n'est pas non plus la fiscalité, qui est déjà confiscatoire. Aider les entreprises en difficulté, c'est bien, mais, pour libérer l'économie, libérez les commerçants, monsieur le ministre, tous les commerçants ! Alors que la Banque de France et l'Insee annoncent la destruction de 800 000 emplois en 2020 et un taux de chômage de près de 11 % en 2021, ne faites pas le « mariole », comme on le dit chez moi, ne parlez pas de relance. Contentez-vous plutôt de mettre en place une politique de grand sauvetage de l'économie française, si vous ne voulez pas que les Français subissent, en plus du grand remplacement, le grand effondrement

Quelques jours avant le coup d'envoi du marathon budgétaire, ce quatrième PLFR fait un peu figure d'échauffement, mais il conclut surtout un exercice budgétaire sans précédent. Avant de vous livrer quelques observations sur le caractère proprement extraordinaire de cette situation, je souhaite d'abord revenir sur son caractère très ordinaire. En effet, ce PLFR remplit aussi la mission ordinaire d'un collectif budgétaire de fin de gestion. Comme lors des années précédentes, le Gouvernement n'a pris aucun décret d'avance et ne propose aucune réforme fiscale. Je tiens à le saluer, car ce n'est pas parce que les temps sont durs que nous devons nous arranger avec la discipline budgétaire, bien au contraire. Cette rigueur renforce la lisibilité et la transparence du travail du Parlement. Alors que notre société est rongée par la défiance et le complotisme, souligner cette rigueur n'est pas pécher par excès de zèle, et pour cause : dans le contexte de crise que nous connaissons, tous nos efforts doivent viser à créer de la confiance, la confiance, qui est le carburant de l'économie. La situation des finances publiques que ce PLFR entérine est catastrophique. En moins d'un an, notre taux d'endettement aura bondi de vingt points. La dépense publique représente désormais près des deux tiers de la richesse nationale, connaissons une récession à deux chiffres : cela a de quoi donner le vertige. Dans ce contexte, nous ne pouvons maintenir la confiance qu'à deux conditions : d'une part, en préservant le tissu économique afin de ménager notre capacité de rebond

En tout, ce sont donc près de 20 milliards d'euros que nous injectons de nouveau dans l'économie afin d'éviter que le virus ne tue aussi nos entreprises Je ne relancerai pas aujourd'hui les polémiques sur l'ouverture des commerces. Nous savons tous, ici, la colère des commerçants et nous la comprenons. Pour rester cohérentes avec ces mesures sanitaires lourdes, monsieur le ministre, les mesures économiques doivent être à la hauteur des restrictions imposées et de leur impact- nous y reviendrons lors de l'examen du projet de loi de finances. finances. Les commerçants, plus généralement l'ensemble des entrepreneurs, voudraient avoir davantage de visibilité. C'est malheureusement impossible, car les mesures sanitaires ne peuvent être actualisées et adaptées que sur des périodes courtes de deux à trois semaines,

pour les acteurs de terrain. Ils lui préfèrent, pour l'heure, les mesures d'urgence en euros sonnants et trébuchants : un tiens vaut toujours mieux que deux tu l'auras ! Aussi, au-delà des discussions que nous aurons sur le bon calibrage de ces mesures, je crois que le message que nous envoyons est clair et cohérent avec les mesures prises depuis le début de la crise : la santé prime, « quoi qu'il en coûte ». C'est pourquoi le groupe Les Indépendants approuve ce PLFR, qui compensera en partie les dégâts du reconfinement. À mes yeux, son principal intérêt réside dans ce qu'il nous permet de préparer la reprise et, donc, de bâtir la confiance dans l'économie. Sans entreprise, pas de reprise ; sans reprise, pas de croissance ; sans croissance, pas de confiance. Pour conclure, mes chers collègues, je souhaite m'attarder sur cette notion de confiance et sur celle de dette qui la menace dangereusement. Certes, nous pouvons nous réjouir que la signature de la France continue d'inspirer la confiance. Le contexte international nous est encore favorable, de même que la politique de la Banque centrale européenne (BCE). Cependant, comme notre rapporteur général l'a souligné, nous devrons attendre plusieurs années avant d'espérer ramener notre taux d'endettement autour de 100 % du PIB. Or il y a quelques mois seulement, le Sénat s'alarmait à juste titre d'un taux aussi élevé. Si nous voulons vraiment nous convaincre qu'il n'y a pas d'argent « magique », alors nous devons très rapidement changer de braquet et réduire drastiquement les dépenses publiques. Il y va de la soutenabilité de notre économie. La parole est à Mme

Ce PLFR n'est pas à la hauteur pour la culture ni pour les petits commerces. Alors que les géants de la distribution, les hypermarchés et la vente en ligne sont les grands gagnants de la crise, vous ne leur demandez rien. Ce projet de loi de finances rectificative n'est pas à la hauteur pour les quartiers populaires. Ce week-end, cent dix maires des villes de banlieue vous le disaient : « En En dépit des alertes, les villes et quartiers populaires restent un angle mort du plan de relance : aucune mesure ambitieuse n'a été prise pour répondre à la détresse sociale et économique qui frappe nos communes. » Pourtant, les « premiers de corvée ceux qui sont en première ligne dans cette crise et qui sont aussi les plus touchés par cette maladie, vivent, pour un grand nombre d'entre eux, dans ces villes et quartiers populaires. Ce projet de loi de finances rectificative n'est pas à la hauteur non plus en matière de logement d'urgence ni de logement social. Il n'est pas à la hauteur pour aider les plus précaires et les publics vulnérables, qui basculent trop nombreux dans la pauvreté. Sur les 20 milliards d'euros d'aides prévus, seul 1 milliard d'euros l'est pour les plus pauvres, soit 5 % des mesures d'urgence, presque rien pour les associations qui les accompagnent et pas assez pour les collectivités qui essaient de faire face mais qui sont dépassées.

je perçois des arrière-pensées, que je qualifierais d'assez sombres et que je ne vois nulle part démenties. Pendant cette crise, vous organisez le transfert de la dette publique vers les comptes sociaux. sociaux. Pourquoi l'assurance chômage finance-t-elle un tiers de la dépense exceptionnelle du chômage partiel, pourtant décidé par l'État ? Quelle réforme de l'assurance chômage devons-nous craindre ? Par ailleurs, en quoi la réforme des retraites devrait-elle participer à payer la dette covid ? Vous nous promettiez qu'avec réforme cette personne n'y perdrait ; or M. Le Maire nous indique que c'est grâce à elle que nous allons réaliser des économies.

et en profiter pour baisser les dépenses publiques, qui ont pourtant un rôle d'amortisseur social. Enfin, vous n'êtes pas à la hauteur de la crise climatique ni de la soif de justice sociale, pourtant tellement forte dans notre pays. Les milliards que vous déversez ne sont soumis à aucune condition, ni sociale ni environnementale. Ils ne sont ciblés ni vers les énergies renouvelables, ni vers les infrastructures de transport, ni vers la réduction des gaz à effet de serre, ni vers le respect du droit du travail et de l'égalité femmes-hommes. Il est

Conditionnez les aides à l'interdiction de verser des dividendes, à des actions vigoureuses pour sauver le climat ou pour réduire les écarts salariaux, par exemple. Que vous le vouliez ou non, la crise écologique et là ; la crise sociale aussi. Organisons la transition vers un autre modèle de développement, ou la bascule sera brutale. sera brutale. Quand nous vous disons « transition énergétique », vous répondez : « soutien aux dépenses polluantes », « refus de la conditionnalité des aides ». Quand nous vous disons « justice sociale », vous répondez par des mesures trop faibles pour aider les plus précaires. nous vous disons « démocratie », vous répondez par des décisions prises en conseil de défense dans la plus grande opacité. Nous devons changer de direction. C'est pourquoi le groupe Écologiste -Solidarité et Territoires, composé d'élus EELV, Générations.s, d'élus de nos territoires, sera là pour proposer un autre chemin

C'est la quatrième fois que nous nous réunissons cette année pour voter un nouveau budget rectificatif. Fidèles à cette maxime, c'est la quatrième fois que nous ajustons les prévisions de la loi de finances initiale et que nous renforçons le soutien de l'État à une économie fortement éprouvée. S'il y a bien une chose que nous avons apprise au cours de ces longs mois de pandémie, c'est qu'il n'y a pas de bonne prévision en temps de crise- un simple coup d'oeil à l'article liminaire suffit à nous en convaincre. nous comprenons également que l'essentiel est ailleurs et qu'une bonne politique d'urgence est une politique qui soutient massivement l'économie et fait en sorte de préserver ce qui doit être préservé pour que, à l'issue de la crise, le pays soit prêt pour la reprise. Les prévisions de ce PLFR 4 sont plus sombres que celles que le Gouvernement avait communiquées il y a quelques semaines, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2021, mais il faut reconnaître qu'elles sont meilleures que celles que nous avions anticipées lors de la discussion du PLFR 3. La résilience de notre économie et de nos concitoyens nous a permis de connaître un rebond inédit de 18 % au troisième trimestre. Notre économie semble prête à repartir au moindre signe d'accalmie, mais, pour l'heure, reconnaissons que la crise sanitaire dicte encore le tempo de la reprise. que le Gouvernement nous a présenté un quatrième budget rectificatif, qui apporte un soutien inédit de 20 milliards d'euros à notre économie et à nos concitoyens ayant le plus souffert de la crise : 20 milliards d'euros ! Dans le tourbillon des chiffres qui s'amoncellent depuis le début de cette crise, on finirait presque par en oublier l'ampleur : 20 milliards d'euros de crédits nouveaux pour faire face à la seconde vague ; 20 milliards qui s'ajoutent aux 66 milliards d'euros déjà dépensés depuis le début de la crise.

dans ce seul budget que l'ensemble des crédits ouverts depuis le début de la crise. C'est une réponse forte aux inquiétudes de nos entreprises, qui subissent de nouveau de plein fouet les restrictions sanitaires. Ce renforcement inédit permet d'élargir le plafond d'aide à 10 000 euros et le plafond d'emplois à 50 employés pour les entreprises visées par une mesure de fermeture administrative. Pour accompagner les plus fragiles, l'État finance également une nouvelle prime de précarité pour près de 1,1 milliard d'euros. Il finance en outre le renforcement de la prime d'apprentissage, de l'allocation aux adultes handicapés et des allocations d'invalidité à hauteur de 500 millions d'euros. Si l'on nous avait Si l'on nous avait dit en février dernier que le chômage partiel aurait ainsi protégé la moitié des salariés de France, personne ne l'aurait cru. Si l'on nous avait dit que l'État consentirait un effort de 6 milliards d'euros par mois pour accompagner les entreprises en difficulté au seul titre du fonds de solidarité, personne ne l'aurait cru. l'on nous avait dit, enfin, que les aides aux plus précaires auraient bénéficié de plus de 1 milliard d'euros de crédits nouveaux pour la fin de l'année, personne ne l'aurait cru. Bien entendu, il y aura des débats ; c'est l'honneur de notre assemblée, car c'est ainsi que nous pouvons ajuster les dispositifs présentés par le Gouvernement et que nous, parlementaires, adaptons la loi aux réalités de nos territoires. Mais je crois que personne, ici, ne remettra en question l'ambition de ce PLFR 4 ni l'ampleur des moyens déployés. bien sûr, des points à compléter. Je m'inquiète, par exemple, pour l'avenir des entreprises de loisirs, qui sont particulièrement touchées et qui ont, depuis le début de la crise, payé le plus lourd tribut à notre politique de prévention. ouvert une enveloppe de 300 millions d'euros destinée à aider le secteur de la culture et du sport, enveloppe dont ces entreprises pourront sans doute bénéficier. Certes, elles seront éligibles au dispositif de droit commun, à commencer par le fonds de solidarité, mais nous attendons encore des précisions quant au soutien que le Gouvernement compte leur apporter. Aujourd'hui plus encore qu'au début de cette crise, nous constatons les effets à long terme de la pandémie sur nos proches, dans nos territoires et dans la société tout entière. Notre responsabilité politique doit être à la hauteur de cet enjeu. Je crois que nous l'avons tous compris, car c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Une nouvelle fois, laissons de côté nos dissensions, nos oppositions politiciennes, et soyons unis pour faire face à l'urgence

Toutefois, c'est aussi à ce moment-là que les contaminations ont commencé à reprendre, avec la liberté retrouvée, mais avec une vigilance que l'on sait désormais insuffisante, car trop rapidement relâchée. Nous nous trouvons donc, une nouvelle fois, en ce mois de novembre, dans une zone de récession et de fortes turbulences. À ce rythme, il devient parfois difficile de suivre l'évolution des prévisions macroéconomiques,

le troisième PLFR, qui a été examiné et adopté en juillet dernier, faisait déjà figure de « pré-PLF », avec plus de mille amendements déposés dans cette assemblée. Ce quatrième projet de budget rectificatif ne modifie pas sensiblement le montant du déficit de 2020, déjà abyssal, il est vrai. Il prévoit des mesures budgétaires complémentaires, ainsi que des ajustements. Les prévisions sont plus pessimistes que dans le PLF 2021, alors qu'on aurait pu espérer une fin d'année moins défavorable.

rehausse de plus de 1 000 ETP le plafond d'effectifs des opérateurs de l'État, en particulier ceux de Pôle emploi. En effet, le service public de l'emploi est déjà et risque d'être de plus en plus sollicité dans les semaines et les mois qui viennent, en raison de la hausse inéluctable du chômage. La « bonne nouvelle » de ce PLFR, c'est que la vingtaine de milliards d'euros de nouvelles dépenses qui sont engagées pour financer le plan d'urgence sera compensée par des recettes supplémentaires, notamment les rentrées fiscales enregistrées pendant l'été.

si un rebond économique devrait avoir lieu en 2021, l'expérience de cette deuxième vague démontre que, tant qu'une solution durable- vaccin ou autre -n'aura pas été trouvée contre l'épidémie, nous ne serons pas à l'abri de nouvelles recrudescences des contaminations et de nouvelles restrictions pour y faire face.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre débat intervient au lendemain d'une annonce très inquiétante faite par la Fondation Abbé Pierre : le nombre de personnes sans logement dans ce pays approche les 300 000. Ces nouvelles viennent quelques jours après la publication du rapport alarmant du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France : pauvreté et inégalités ont augmenté depuis dix ans dans notre pays, de façon continue, et l'on annonce que la France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020. Mes chers collègues, vivons-nous bien dans la sixième puissance économique du monde ? Ce projet de loi de finances rectificative, quatrième du nom pour cette année, répond-il à ces enjeux ? Nous répondrons par la négative, à l'examen des chiffres. En effet, vous accordez une aumône de 150 euros, pendant un mois seulement, aux chômeurs en fin de droits, aux étudiants boursiers et aux bénéficiaires de l'APL. L'association ATD Quart Monde dénonce « des mesures pansement, déconnectées de la vie des gens, loin d'être à la hauteur de la situation ». Est-ce bien crédible, au moment où chaque jour sont annoncés des plans de licenciements, qui vont faire basculer dans la précarité des milliers de salariés et leurs familles ? Nous sommes bien loin du « quoi qu'il en coûte » présidentiel. Le traitement des inégalités et de la pauvreté est, selon nous, le principal échec de ce projet de loi de finances rectificative. Notre groupe propose, au travers de ses amendements, des mesures concrètes pour répondre à ce défi social urgent : revalorisation et extension du revenu de solidarité active (RSA), augmentation des bourses étudiantes et aide au logement pour les plus démunis. Il est temps de mettre à contribution ceux qui n'ont pas été au rendez-vous de la solidarité, et d'autres qui parviennent même à sortir gagnants de la pandémie qui nous frappe. Il s'agit, par exemple, des compagnies d'assurances, qui disposent d'un confortable matelas de 100 milliards d'euros de

Ces groupes payent trois fois moins d'impôts que le libraire du quartier. Ainsi, quand Google paye son impôt, c'est au terme d'une bataille judiciaire de plusieurs années. a ainsi réglé, il y a quelques mois, une somme de 500 millions d'euros, plus 400 millions de pénalités, mais ce chèque venait solder un litige qui portait sur 7 milliards d'euros d'impôts éludés par Google pendant dix ans. Le fisc s'est donc assis sur 6 milliards d'euros ... Autrement dit, « fraudez, fraudez, il en restera toujours quelque chose ! » Le constat que nous pouvons faire à l'occasion de ce PLFR 4 est le suivant le Gouvernement, même en pleine pandémie, ne remet pas en cause ses fondamentaux. Il est hors de question de solliciter les plus hauts revenus et les dividendes par l'impôt ; et puis l'on entend discrètement revenir à l'ordre du jour le néfaste projet de réforme des retraites. réforme structurelle fait partie de celles qu'exigent l'Union européenne, la Banque centrale européenne et les marchés financiers, ceux-là mêmes que vous allez encore favoriser, car, en ne mettant pas à contribution les dividendes, les grosses fortunes et les patrimoines, vous faites le choix d'avoir recours à la dette. Pour dire les choses plus trivialement, « c'est celui qui paye les musiciens qui choisit la musique » ! Or cette dette inquiète nos concitoyens. Chacun et chacune s'interroge : qui va la payer ? M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, a apporté la réponse, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale : « Cette dette, je tiens à le redire, elle devra être remboursée le moment venu par la croissance, par un effort de responsabilité en matière de dépenses publiques et par des réformes structurelles, dont la réforme des retraites. » Ce projet de loi de finances rectificative ne prend pas le chemin de la nécessaire solidarité. Il ne prend pas en compte, selon nous, la gravité de la crise sociale qui est renonce à solliciter les très hauts revenus et à taxer les dividendes. Nous défendrons nos propositions de justice sociale et fiscale, durant le débat de ce jour. En l'état, ce PLFR 4 n'offre pas de vraies réponses à la situation de notre société. Le groupe CRCE ne pourra y apporter son soutien.

si nous sommes réunis, cet après-midi, c'est bien parce qu'une seconde période de confinement a été décidée, durant cette année 2020, dans notre pays. Or qui dit confinement,

les cartes. Nous avons le droit de déplorer le manque d'anticipation, car le conseil scientifique a tiré la sonnette d'alarme dès cet été. Dans son avis du 27 juillet, il prévoyait une croissance exponentielle de la circulation du virus pour le mois d'octobre suivant. Il l'a confirmé en septembre dernier. Pourtant, le Gouvernement a attendu pour agir, a relâché le protocole sanitaire dans les écoles et il a tardé à reconnaître la mise en échec du système de dépistage et de traçage. La conséquence, c'est que vous n'avez pas pu éviter de prendre de nouvelles mesures de confinement très strictes. Lorsqu'on ne donne pas la priorité au sanitaire, il se rappelle de toute façon à vous, encore plus fort. Prises tardivement, les mesures de restriction pèsent aujourd'hui très lourdement sur notre économie. Monsieur le ministre, nous nous retrouvons donc avec un PLFR 4 qui ressemble beaucoup aux trois premiers. Vous avez revu votre copie et vous évaluez désormais à 11 % la chute du PIB cette année, le déficit à 11,3 % et la dette publique à 120 %. Ces chiffres impressionnants, vous n'en êtes bien sûr pas entièrement responsable, car la pandémie est mondiale, mais vous auriez pu atténuer cet échec par une meilleure organisation sanitaire, comme l'Allemagne a réussi à le faire. Disons-le aussi, ce texte rend caduque toute la politique économique et fiscale menée depuis 2017 au nom de la compétitivité et du fameux « ruissellement

la prise en charge du chômage partiel et le soutien aux entreprises qui doivent réduire ou arrêter leur activité. Toutefois, cela ne suffit pas. Il faudrait que les mesures qui ont été prises soient bien davantage ciblées sur les victimes de ce nouveau choc, sur les entreprises comme sur les Français les plus durement touchés par la crise. À cet égard, votre plan de relance apparaît insuffisant et mal calibré, et vous sous-estimez gravement l'explosion de la pauvreté dans notre pays. Il est encore temps d'écouter la représentation nationale et de faire évoluer votre projet. Sur plus de 500 amendements présentés à l'Assemblée nationale, neuf seulement ont été adoptés, dont un seul n'émanait pas du Gouvernement.

On soutiendrait la demande, et la mesure serait efficace économiquement et socialement. Nous vous proposons aussi la hausse de 100 euros par mois du RSA, pour les trois derniers mois de l'année, et son extension aux jeunes en situation de précarité. Très bien ! En effet, comment accepter que la crise sacrifie ainsi une génération ? Le Secours catholique estime que la barre des 10 millions de pauvres en France sera dépassée cette année. Toutes les associations et les syndicats vous demandent d'agir davantage. Entendez-les ! Écoutez l'économiste Esther Duflo quand elle dit : « Il faudrait revaloriser le RSA beaucoup plus largement, s'appuyer sur l'APL pour donner un revenu aux jeunes, en tout cas pour les mois à venir. D'autant que des minima sociaux plus élevés accroissent la demande et soutiennent la reprise de l'activité : dans une telle période de récession, ils ne sont en rien un frein à l'emploi, toutes les études le démontrent. Nous vous proposons également d'accroître le soutien à l'aide alimentaire, car les associations voient les files d'attente s'allonger sans cesse. Elles tirent le signal d'alarme, si bien qu'il est indispensable de les aider davantage dès cette fin d'année, et bien sûr ensuite dans la loi de finances pour 2021. Enfin, nous vous proposons de prendre en charge les dépenses d'achat des masques, puisqu'ils sont désormais obligatoires, notamment en milieu scolaire. Pourquoi le Gouvernement s'entête-t-il à refuser une telle mesure de bon sens ?

dernier volet d'une regrettable série, tant nous aurions préféré ne pas avoir à les voter. Cependant, la pandémie qui frappe le monde est venue bousculer l'année 2020, en emportant avec elle des vies et des modes de vie, et en ébranlant notre pays déjà en peine dans son dynamisme économique. que jamais nous n'aurions pensé vivre une telle situation, jusque-là inédite, c'est toute notre nation, ordinairement vivante, vaillante et audacieuse qui a dû se résoudre à s'enfermer, entraînant par là même l'arrêt quasi complet de notre économie. Trois mois durant, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, des entreprises ont souffert, parfois même jusqu'à en mourir, car elles n'avaient plus les rentrées ou la trésorerie suffisantes pour pouvoir honorer leurs engagements et leurs charges.

voilà maintenant plus de deux semaines que nous sommes confinés et que, sans consultation ni concertation, vous avez décidé de stopper notre économie. Même s'il existe bel et bien un virus qui cause énormément de dégâts dans notre pays, ce que nul ne peut nier, il existe également une situation que le Gouvernement a créée par son manque d'anticipation et qui va, elle aussi, causer de nombreux dégâts.

L'économie est sacrifiée au profit de la santé, mais rappelons-nous que l'économie c'est précisément la santé et l'assurance d'éviter des cas tragiques de détresse psychologique, qui poussent parfois certains à commettre l'irréparable.

Ce confinement est un désastre, et les Français ne comprennent pas son manque de cohérence. On laisse ouvertes les grandes surfaces, mais en même temps on ferme les petits commerces. On ferme les restaurants de campagne, alors qu'ils respectent les distances de sécurité, mais en même temps on laisse ouverts les restaurants d'entreprise ou les cantines à grande fréquentation.

stupéfait d'entendre, le week-end dernier, les absurdités de la ministre du travail ? Elle demande aux entreprises des stations de ski d'embaucher quelque 120 000 saisonniers, puis de les mettre au chômage partiel, payé par l'État, si le confinement dure

Toutes ces entreprises qui concourent ordinairement massivement à la richesse de l'État sont aujourd'hui à l'arrêt. Par un effet pervers de votre politique, ce sont ceux qui y contribuent le moins qui en perçoivent désormais la majorité des bénéfices. Il s'agit, vous l'aurez compris, des géants Gafam que vous aviez promis de taxer, mais qui ne contribuent finalement que marginalement à la richesse de notre pays, tout en détruisant des emplois.

qui devrait par ailleurs chuter de 11 % à cause du confinement ! Vous venez aujourd'hui nous demander la bagatelle de 20 milliards d'euros. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, ce PLFR est loin de nous satisfaire. Cependant, même si c'est à contrecoeur, nous allons voter ce budget, car il est indispensable de venir en aide à nos entreprises, maintenant que le Gouvernement les a mises dans cette triste situation. Prenez donc ce vote non pour un chèque en blanc, mais plutôt comme un pansement que nous offrons à ceux qui en ont aujourd'hui gravement besoin. Nous demeurons opposés à vos prises de décision dans cette gestion de l'épidémie : il faut que vous le sachiez. Même s'il est déjà tard, il n'est pas encore trop tard. Écoutez les Français ; plutôt que de les mettre sous perfusion, permettez-leur simplement de travailler

Bien que nous ne contestions pas la nécessité d'agir en responsabilité, afin d'endiguer la crise sanitaire, nous nous interrogeons sur l'équité de vos décisions. Les grandes surfaces sont grandes ouvertes, et elles captent toute la clientèle dans un espace clos et concentré. Les petits et moyens commerces sont fermés. Pourtant, ils sont en mesure d'assurer de manière responsable un protocole sanitaire strict, tout en poursuivant leur activité. Le choix a été de sacrifier les petits au profit des gros. Or les gros, ce sont non pas seulement les grandes surfaces, mais aussi les géants du e-commerce ; je ne vous apprends rien. Alors que le pays était à l'arrêt entre mars et avril derniers, le commerce en ligne a généré 44,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année 2020, soit une hausse de 13 % par rapport au premier semestre de l'année 2019. Au total, près de 50 % de la population française a consulté des sites de vente en ligne sur la même période. Alors que vous connaissez ces données, comment ne voyez-vous pas le danger qui se profile pour nos petits commerçants à l'approche de Noël ? de Noël ? Ils sont directement ou indirectement touchés par cette concurrence déloyale. Je pense par exemple aux producteurs de fleurs de notre pays, qui ont vu toutes leurs perspectives économiques s'effondrer après la fermeture des fleuristes.

Surtout, j'espère que vous accorderez une place plus importante à l'accompagnement financier de nos petits commerçants, qui assurent à eux seuls la vitalité de nos territoires et perpétuent un savoir-faire français. Ces commerçants ne sont malheureusement pas les seuls oubliés de ce texte. En ces temps de pandémie, où le maître mot est « restez chez vous, sauvez des vies », il semble indispensable de garantir un « chez-soi » au plus grand nombre et, particulièrement, aux plus vulnérables.

il apparaît primordial de protéger les plus précaires. Avec l'article 1, vous semblez emprunter un tout autre chemin. Aussi, nous espérons que vous adopterez l'amendement que nous proposons, afin de supprimer cet article anachronique. Si cela vous semble irréaliste, gardez en mémoire que tous les voyants sont au rouge. J'en veux pour preuve le rapport du Secours catholique paru la semaine dernière, qui prévoit une hausse significative des défauts de paiement en matière locative et l'apparition de 10 millions de pauvres dans notre pays. Ce constat devrait nous amener collectivement à redéfinir les priorités de ce plan d'aide. En effet, grands absents de votre plan de relance, les plus précaires paient un lourd tribut dans cette crise. Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui avait été décidé lors de la crise financière de 2008 : à l'époque, les mesures de solidarité correspondaient à 8,3 % du plan de relance, tandis qu'elles ne représentent plus que

En conclusion, je précise que ce texte traduit votre philosophie habituelle : un soutien massif et aveugle aux grosses entités, un service minimum pour les petits et moyens de ce pays, et une aide dérisoire pour les plus précaires. Dans ces conditions nous ne pourrons pas voter ce texte en l'état.

C'était le cas des précédents mais, cette fois, il faut boucler l'année et donc « viser juste » en termes de crédits. À cela s'ajoute un reconfinement dont la durée est hypothétique, mais qui devrait malheureusement s'accroître.

à lire dans le marc de café : les données des cartes bleues, celles de la mobilité ou de la consommation d'électricité. Il faut évaluer la situation au fur et à mesure ; or elle est mouvante.

dépenser plus pour faire face à la situation sociale et économique qui se présente à nous, maintenir l'emploi et le tissu productif. Toutes ces questions sont devant nous.

de la crise actuelle sur les plus fragiles et les personnes en situation précaire est majeur. Des mesures ont été prises, mais il faudra sans doute les amplifier. C'est un sujet de solidarité, de cohésion sociale, mais c'est aussi un enjeu pour la demande de demain. Abordant ces questions, je me dois de souligner que le vote que nous allons exprimer ne vaut pas quitus. La situation sanitaire et son impact économique commandent. Sur ce plan, nous avons le sentiment que le Gouvernement a vu, comme d'autres, la situation lui échapper. Monsieur le ministre, par souci de responsabilité, le groupe UC votera, au bénéfice de ces observations, ce PLFR 4 amendé par le Sénat. Nous serons Nous serons vigilants pour faire face à la situation exceptionnelle à laquelle nos compatriotes sont confrontés.

s'il n'y a pas de chômage partiel, il y a du chômage tout court ; s'il y a du chômage tout court, l'Unédic le finance à 100 %. Notre choix a donc été de mettre en place un système de protection de l'emploi et des compétences par le chômage partiel à un niveau qui n'avait jamais été atteint dans notre pays. En effet, nous avons gardé en tête le

prévoit des lignes de crédits particulièrement importantes pour les secteurs de la culture et du sport, y compris en mobilisant des dépenses accidentelles et imprévues. Je voudrais aussi rassurer le président Requier et, à travers lui, l'ensemble de celles et ceux qui s'inquiéteraient du niveau suffisant ou insuffisant des crédits que nous ouvrons pour faire face à la crise. J'ai déjà eu l'occasion de le dire rapidement dans mon propos liminaire

qui nous séparent de la fin de l'année. Nous avons préféré, pour reprendre les mots utilisés par plusieurs d'entre vous, faire preuve de prudence en la matière. M. le rapporteur général l'a souligné et je l'en remercie, nous préférons avoir de quoi voir venir : si les crédits n'étaient pas consommés, parce que l'activité est plus forte que prévu, ce serait une bonne nouvelle que nous serons les uns et les autres prêts à partager.

à la fois de l'évolution de la situation et d'un certain formalisme, qui tient aux dates de saisine et de remise des avis du Haut Conseil des finances publiques. Cependant, c'est la seule solution que nous avons trouvée pour garantir que, à la fin de l'année 2020,

qu'elle estimait que notre hypothèse d'une baisse d'activité de 20 % en novembre était supérieure à sa propre lecture de la situation, puisqu'elle l'évalue à 12 %. Mais, en la matière, comme depuis le début de cette crise et comme depuis plusieurs années,

d'un exercice particulier : le présent PLFR comporte à la fois le schéma de fin de gestion d'un projet de loi de finances que beaucoup d'entre vous ont certainement rejeté au début de l'année,

entend parfaitement celles et ceux qui, parmi vous, disent voter ce texte pour répondre à l'urgence, sans partager les orientations fiscales ou budgétaires du Gouvernement. Nous aurons l'occasion d'en

entreprises : subir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % ; avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, soit le seuil maximal retenu pour définir une PME. J'ajoute que les reports des échéances sociales et fiscales ont été parfaitement bien perçus

et ne prendrait pas en compte la diversité des situations des entreprises répondant aux critères. En effet, l'amendement vise à la fois les cotisations sociales et les impôts directs, dont des impôts locaux, pour un enjeu financier considérable. Quel est l'avis du Gouvernement

une fois n'est pas coutume, je vais m'associer à la majorité présidentielle et défendre l'esprit de l'amendement voté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de la députée Aude Amadou, par ailleurs sportive professionnelle et

il n'y a pas que ces professionnels dans le monde du haut niveau. Il est important pour de nombreux et de nombreuses athlètes de haut niveau d'être protégés.

j'y souscris, j'y reviendrai -, je note que le Gouvernement applique cette règle quand il s'agit de ne pas introduire de mesures fiscales concernant les plus aisés de nos concitoyens- mais c'est un autre sujet ... En tout cas,

quelles solutions, en dehors du groupe de travail que vous avez évoqué, allez-vous proposer spécifiquement sur ce sujet pour améliorer la situation de nos sportifs, et surtout de nos sportives ? Entendez-vous déposer un amendement dans le cadre du

Il permettait d'apporter une aide non négligeable aux clubs et avait également pour objet de renforcer l'attractivité sportive de notre pays. Le rétablissement de ce DIC est une demande unanime de l'ensemble des acteurs du sport professionnel. Quand je parle de sport professionnel, je ne pense pas uniquement au foot masculin, mais je parle également du hockey sur glace, du handball, du rugby, du basket-ball, du volley-ball masculins et surtout féminins. Je tiens à rappeler ici que la situation économique des clubs de sport professionnels est aujourd'hui très compliquée du fait de la situation sanitaire. Un dispositif, qui devait devenir un nouveau droit à l'image des

J'entends aujourd'hui l'opposition du rapporteur général et du Gouvernement à cet article 1 A, mais nous devons avoir des engagements clairs et précis : une simple opposition de principe pour mieux enterrer le dispositif ne suffira pas. Monsieur le ministre, à l'issue d'une rencontre que vous avez eue avec le syndicat Première Ligue il y a trois mois, son président a déclaré : « La discussion avec M. le ministre a été constructive. Nous espérons désormais qu'elle se traduira par des actes concrets dans le plan de relance et dans les textes budgétaires à l'automne. »

soit le Gouvernement, par votre voix, s'engage, non pas à proposer, une simple réunion de travail, mais à présenter rapidement devant le Parlement, lors d'un prochain débat budgétaire, un nouveau dispositif sur lequel nous serions prêts à travailler, et qui devra irriguer l'ensemble du sport professionnel.

je voudrais d'abord souligner- je le dis à l'attention du président Kanner et en écho à ses propos -que nous parlons, s'agissant du dispositif qui a été voté à l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur général et du Gouvernement, mais qui est aussi l'expression d'un vote dans l'hémicycle, l'hémicycle, d'un droit à l'image collective et en aucun cas individuelle. Or la solution pour un bon nombre d'athlètes réside plus certainement dans la réforme et l'amélioration du droit à l'image individuelle que dans le droit à l'image collective, celui-ci se heurtant à plusieurs difficultés.

sur lequel vous aviez une tutelle, puisqu'il était votre secrétaire d'État lorsque vous étiez ministre des sports. Vous connaissez donc parfaitement le dispositif tel qu'il a été conçu. Or ce dispositif fonctionne mal. M. Savin l'a dit, à l'occasion d'une rencontre avec les représentants du syndicat Première Ligue,

et cohabiterait avec un dispositif réintégrant celui de 2010, dont nous connaissons aussi d'expérience ou à la suite des lectures les limites et les lacunes, notamment sur la concentration des bénéfices au profit des clubs les plus fortunés ou les plus favorisés, et des sportifs les plus riches. Il nous faut trouver un système qui soit finalement entre les deux : un dispositif qui ne soit pas le DIC de 2010 avec les défauts, qui avaient été décrits et avaient fait l'objet de multiples rapports, notamment de la Cour des comptes, et un dispositif qui ne soit pas le DIC de 2017, dont nous avons vu

sans rétablir un dispositif dont nous connaissons les limites en termes de coût pour la sécurité sociale et pour l'État, ainsi que d'injustice dans la répartition des sommes, et sans

à la condition que ces sociétés emploient au moins un ou deux salariés à la clôture de l'exercice suivant celui de la souscription.

sera pour certaines d'entre elles impossible à tenir, sauf à engager artificiellement leurs fonds à cet effet, et au péril du devenir de la société, dont l'activité n'aura parfois pas encore pu débuter au 31 décembre 2020. Cet

de passer outre cette pandémie, il serait curieux de ne pas permettre à celles qui ont été mises sur les fonts baptismaux en 2019 de survivre et de prospérer. Elles portent souvent en germe l'avenir de notre économie. Ce sont même souvent des entreprises très novatrices.

Monsieur le ministre,

solliciter la contribution du secteur financier pour les finances publiques, réguler le marché boursier et susciter l'adhésion des autres États membres de l'Union européenne pour une portée plus générale. Nous le savons, les débats s'enlisent et le secteur le secteur financier ne contribue pas beaucoup, en tout cas pas à la hauteur des volumes qu'il brasse chaque année. Par exemple, le plus petit volume d'échanges sur une journée, depuis 2010, a été de 808 millions d'euros,

l'avis de la commission ?

à l'effort de la Nation face à la crise, et ce sans s'attaquer au patrimoine et aux économies de la classe moyenne ou des Français les plus modestes. Nous savons bien que l'assurance vie est un instrument d'épargne très largement répandu.

l'avis de la commission ?

Monsieur le ministre,

des instruments de droit commun et transversaux, que ce soit le chômage partiel, les reports d'échéances de paiement de cotisations et de contributions sociales, ainsi que le fonds de solidarité, dès lors que les critères,

Le secteur de la conchyliculture, s'il était éligible dans les règles communes au secteur agricole, pouvait en bénéficier. Au-delà, nous savons la situation particulière du secteur de la conchyliculture et de la pisciculture. Aussi, dans le cadre du projet

le plus rapidement possible.

j'aimerais une nouvelle fois attirer votre attention sur les contradictions inhérentes à la suppression de la taxe d'habitation pour certaines communautés de communes. En effet, les communautés de communes issues de fusions ont dû mettre en place des mécanismes de lissage des taxes qu'elles prélevaient. Cela supposait des diminutions de taux sur certaines parties du territoire et des augmentations sur d'autres parties, afin d'aboutir à un produit fiscal constant pour la nouvelle communauté, et et ce sans prélèvement supplémentaire sur l'ensemble du territoire. Un tel lissage a nécessairement impliqué une augmentation du taux de la taxe d'habitation sur certaines parties du territoire,

de mettre à la charge des collectivités concernées la partie des dégrèvements de la taxe d'habitation 2020 correspondant à l'augmentation des taux qu'elles auraient décidée entre 2017 et 2019. Sans aucune mesure de différenciation entre les communes, un tel mécanisme apparaît foncièrement injuste et contrevient à l'objectif de cohérence fiscale territoriale et de lissage. Ce PLFR Ce PLFR 4- j'en ai bien conscience -a vocation à se concentrer sur le schéma de fin de gestion et sur les mesures d'urgence liée à la crise. Toutefois, monsieur le ministre, pourriez-vous me préciser vos intentions, afin qu'une solution soit trouvée aux problèmes rencontrés par les EPCI issus de fusions en cours d'intégration fiscale ? Pour eux, le trou dans la raquette qui demeure dans le schéma de compensation est source de profondes injustices. Je suis saisi

La formule est un peu curieuse en droit organique et même en droit constitutionnel. Cette cotisation est en fait un impôt déguisé, une imposition de toute nature. Et l'État propose

Les derniers chiffres sont éloquents. Selon une étude du comité olympique publié la semaine dernière, les pertes se chiffrent au minimum à 376 millions d'euros pour 36 000 clubs de sport amateur. C'est un désastre non seulement économique, mais aussi humain et social. L'Agence nationale du sport a créé cet été un fonds territorial de solidarité visant à soutenir les associations, les acteurs sportifs sur nos territoires, tant sur le volet développement des pratiques que sur le volet haute performance. Ce fonds a été doté initialement de 15 millions d'euros provenant d'un redéploiement de crédits de l'Agence nationale du sport, 8 millions d'euros, et d'un abondement de crédits du ministère des sports, 7 millions d'euros. Le 27 octobre dernier, devant notre commission, votre collègue ministre chargée des sports a annoncé que les demandes pour ce fonds se chiffraient à 21 millions d'euros et qu'elle allait demander 6 millions d'euros supplémentaires.

l'éligibilité au FCTVA à la totalité d'un achat financé pour moitié par un partenaire, en l'occurrence l'État.

les services de l'État devraient procéder dans des temps record au traitement des pièces que les collectivités territoriales pourraient leur transmettre.

je vois mal comment on pourrait articuler la contemporanéisation avec l'automatisation, qui doit enfin être mise en oeuvre, après une si

l'avis du Gouvernement ?

proposons de supprimer les pénalités dues par certaines collectivités dans le cas d'une hausse de la taxe d'habitation entre 2017 et 2019, dans le cadre d'un accord de gouvernance.

Pour autant, l'exercice 2020 ne se traduira pas seulement par la poursuite et l'aboutissement des dispositions introduites en loi de finances pour 2018, dont l'objet est de supprimer la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables.

aux nombreuses situations caractérisées par une substitution de fiscalité communautaire à la fiscalité communale. Ainsi, pour de nombreux EPCI, l'augmentation du taux de taxe d'habitation a eu pour contrepartie une diminution des taux de taxe

être mise à la charge des collectivités territoriales par un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. Vous proposez de supprimer cette reprise lorsqu'elle concerne des ensembles intercommunaux ayant modulé leur taux de taxe d'habitation dans le cadre d'un accord de gouvernance financière.

du pacte de gouvernance ou du pacte financier et fiscal ? Pour cette raison, je sollicite l'avis du Gouvernement.

obligatoire de l'augmentation subie. Au-delà des interrogations sémantiques de M. le rapporteur général, que je partage, vous proposez que l'État vienne compenser ou annuler le prélèvement pour des communes qui, au sein d'une intercommunalité, ont fait le choix de conclure un accord de gouvernance. Vous

Elles sont de différents types : gestion directe de la crise, surcoût des contrats de commande publique, renflouement de structures en difficulté, comme les syndicats de communes, ou dépenses en matière sociale. Leur prise en charge par l'État est très insuffisante, puisque celle-ci se résume à un remboursement à hauteur de 50 % des achats de masques, conditionné à une commande réalisée après le 13 avril. Par ailleurs, le dispositif de compensation des pertes de recettes des collectivités locales, adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2020, ne prévoit pas de compensation des dépenses du bloc communal liées à la crise. Aussi cet amendement vise-t-il à garantir que ces dépenses supplémentaires soient compensées par l'État. Monsieur Bocquet, le

Ce compte, tout en préservant l'orthodoxie comptable et la séparation entre fonctionnement et investissement, permet l'étalement sur cinq ans des dépenses de fonctionnement liées au covid, et donc une forme d'amortissement. Cela nous paraît utile pour la trésorerie des collectivités et pour leurs capacités à préserver le maximum d'épargne de fonctionnement

» entre baisse de leurs recettes et hausse de leurs dépenses. Nous avons pu regarder les récentes évaluations de la Banque Postale, qui sont sans appel.

par une part de TVA, devraient baisser de 15 % en 2020, participant à ce recul. Notre amendement tend à apporter à ces départements un soutien fort face à leur perte de recettes. Nous estimons que les avances remboursables pour compenser les pertes de droits de mutation à titre onéreux sont insuffisantes et ne font que décaler le problème, telle une véritable bombe à retardement. Par ailleurs, les conditions d'éligibilité de ces avances ont rendu cette mesure encore plus décevante, puisque de nombreux départements n'ont pas pu en profiter. À ce stade, je me vois contraint de partager avec vous un constat qui me semble effarant : sur les 2,7 milliards d'euros de crédits débloqués, moins de 500 millions bénéficieront aux départements ! Monsieur le ministre, au lieu d'annuler des crédits, améliorons les compensations aux collectivités ! Nous proposons de remplacer ces avances remboursables par une réelle compensation des pertes

l'avis de la commission ?

Il y aura une régularisation après acompte et les départements seront de nouveau tous interrogés. Je rejoins M. Savoldelli sur un point ; la somme sera très certainement inférieure à ce qui a été provisionné, pour une unique raison : la baisse des DMTO en 2020 est bien moins importante que ce que nous craignions lors de l'examen du PLFR 3. Dans la mesure où il s'agit d'un mécanisme de compensation, si les recettes sont plus importantes que prévu, la compensation baisse au fur et à mesure de l'augmentation

moins d'énergie. Pour cela, elles peuvent se faire financer soit par des subventions publiques, soit par des dispositifs de type certificats d'économie d'énergie (C2E), qui visent cet objectif.

commission ? Actuellement, seules sont amortissables les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'État ou les collectivités publiques. L'extension de cette possibilité aux financements attribués les certificats d'économie d'énergie dépasse le champ de l'article, qui réserve ce bénéfice aux subventions publiques.

dont certains rapports ont pu montrer qu'ils présentaient parfois un caractère inflationniste. Au-delà de l'extension d'un mécanisme d'étalement réservé aux subventions publiques à un financement privé- même s'ils sont émis par l'État,

les C2E participent de l'action publique. Le fait de ne pas pouvoir les intégrer dans l'étalement des amortissements ne va pas dans le bon sens.

est une anomalie qui doit être rectifiée. À mon sens, le Sénat pourrait contribuer à cette rectification, dans l'intérêt général.

national si l'on ne renégocie pas les conventions fiscales internationales avec nos partenaires. Vous l'avez évoqué, cela relève de négociations au sein de l'OCDE.

leur faveur une contribution exceptionnelle de la part des grandes surfaces et des plateformes de e-commerce, comme Amazon. Ces établissements ont été moins touchés par la crise que les commerces de proximité ; ce n'est rien de le dire le dire ! Les grandes et moyennes surfaces ont pu rester ouvertes malgré les confinements. Au moment du deuxième confinement, pendant que les commerces de proximité étaient fermés, elles ont pu bénéficier des atermoiements du Gouvernement sur la définition des produits de première nécessité. nécessité. Les plateformes de e-commerce peuvent être considérées comme les grandes gagnantes de la crise sanitaire. Alors que le pays était à l'arrêt entre mars et avril 2020, leur activité économique n'a pas cessé. Le commerce en ligne a généré 44,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année 2020, soit une hausse de 13 % par rapport au premier semestre de l'année 2019.

de la suite éventuelle du projet de loi de finances rectificative pour 2020, mardi 17 novembre, le soir, après l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Acte est donné de cette demande. Nous pourrions d'ores et déjà ouvrir les séances de cette nuit et, éventuellement, de celle de demain pour l'examen de ce texte. Enfin, dans le cas où nous n'aurions pas terminé l'examen du projet de loi de finances rectificative cette nuit, nous pourrions fixer l'heure de reprise de demain soir Dans le cas contraire, nous reprendrions nos travaux à vingt et une heures trente pour l'examen du seul projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Y-a-t-il des observations ?